La séance est ouverte.

compétition internationale réunissant les meilleures formations de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, la CONCACAF. Vous le savez, cette sélection est gérée par la Ligue de football de la Guyane, laquelle est placée sous l'égide de la Fédération française de football. En sa qualité de membre de la CONCACAF, elle peut donc prendre part à la Gold Cup après accord express de la Fédération française de football. Au cours de cette compétition, la Ligue de la Guyane a été sanctionnée pour avoir aligné un ex-international français.

à un match international avec une formation d'un pays membre de la FIFA de jouer avec la formation d'un autre membre. Madame la ministre, au-delà de cette sanction juridiquement contestable, je souhaite appeler votre attention sur la confusion induite par le statut hybride réservé à la sélection de Guyane et, plus largement, à toutes les sélections régionales d'outre-mer désireuses de participer aux compétitions dans leur bassin géographique. Pour rappel, la question s'était déjà posée en 2007 lors de cette même compétition. Un joueur guadeloupéen, Jocelyn Angloma, pourtant ex-international français, avait alors été autorisé à prendre part aux matchs de la sélection de la Guadeloupe. Devant cette situation qui voit une autorisation devenir une interdiction d'une édition à l'autre, quelles actions le Gouvernement peut-il engager pour aider les sélections régionales d'outre-mer à participer à cette manifestation sportive internationale dans de meilleures conditions ? Êtes-vous prête à engager une large réflexion avec la FFF et les sélections régionales sur l'élaboration d'un statut adapté permettant de mieux sécuriser la participation de ces dernières aux compétitions internationales ?

et évolué dans le bassin caribéen. Permettez-moi de rappeler quelques éléments permettant d'éclairer la situation, mais surtout le statut de la ligue de football de Guyane et son rattachement comme membre de la CONCACAF. Pour les départements et régions d'outre-mer, il convient de distinguer l'affiliation aux instances sportives internationales de zone de l'affiliation aux fédérations sportives internationales. L'affiliation des comités régionaux, départementaux ou clubs d'outre-mer à des instances sportives regroupant plusieurs pays d'une même zone géographique et organisant des compétitions entre ces territoires est prévue, sous certaines conditions, dans le code du sport. Sur le plan sportif, cela présente l'avantage d'étoffer le calendrier de compétitions des sportifs concernés et de disposer d'une concurrence de qualité en limitant la contrainte de déplacement. Toutefois, il me semble important de souligner que les fédérations sportives internationales ont vocation à fédérer les associations qui assurent le développement et l'organisation de la discipline concernée dans un pays. Pour un même pays, il ne peut y avoir deux associations affiliées à une fédération internationale. telle situation poserait en effet deux difficultés : d'une part, l'équipe de France pourrait être amenée à affronter une sélection régionale française dans une compétition mondiale ; d'autre part, les sélections nationales pourraient se voir privées de certains talents ultramarins qui préféreraient participer aux compétitions mondiales au sein de leur équipe régionale. Au regard des dispositions du code du sport, les ligues de Martinique, de la Guadeloupe et de Guyane et le district de Saint-Martin ne peuvent adhérer directement à la FIFA. Pour faire évoluer le profil des joueurs sélectionnables au sein des équipes régionales, il conviendrait de modifier les statuts de la FIFA.

pour restreindre son avancée sur le territoire français, plusieurs arbustes ont été de nouveau identifiés comme porteurs de la bactérie, notamment dans les communes d'Antibes et de Saint-Laurent-du-Var, au mois de juillet dernier. Afin de lutter contre la propagation, une délimitation par zone dite infectée de cent mètres autour des végétaux contaminés est imposée et des arrachages sont pratiqués en cas de contamination avancée. avancée. Toutefois, les résultats n'ont pas été concluants : la bactérie s'est propagée et des zones « tampons » de dix kilomètres autour du foyer de la zone infectée sont même aujourd'hui délimitées. Cette année, les arbustes atteints ont été détectés dans le cadre de la surveillance renforcée des zones infectées et, géographiquement, à l'intérieur même de ces zones tampons. Ainsi, depuis le mois de juillet 2015, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on dénombre 3 802 prélèvements analysés, 228 espèces végétales sensibles à la bactérie et 67 arbustes contaminés. contaminés. Les pépiniéristes des Alpes-Maritimes sont inquiets. En effet, leur activité économique est particulièrement frappée, avec des effets indéniables sur l'emploi.

Les nouveaux cas détectés portent à vingt et un le nombre de foyers découverts en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont dix-sept dans le seul département des Alpes-Maritimes. Les protocoles européens d'endiguement et leur application dans nos territoires ne suffisent plus. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie du Gouvernement pour renforcer la lutte contre cette bactérie classée comme l'une « l'une des plus dangereuses au monde pour les plantes » par les autorités européennes et tristement surnommée l'« ebola de l'olivier » en Italie,

végétales et touche directement les agriculteurs, les pépiniéristes, les jardiniers amateurs, les espaces verts et naturels. Elle peut causer des dépérissements très importants. C'est dans votre département. Malheureusement, il n'existe pas de moyen curatif aujourd'hui. Les mesures à prendre en cas d'apparition de foyer sont définies dans le règlement européen. Les services de l'État notifient la destruction des végétaux sensibles dans la limite de cent mètres autour du végétal contaminé et organisent une surveillance intensive dans un rayon de dix les mouvements de végétaux susceptibles d'avoir été contaminés par cette bactérie, dits « végétaux spécifiés », sont strictement encadrés pour éviter la dispersion dans des zones réputées indemnes.

de prendre en compte l'expérience acquise et la grande diversité de situations sur le territoire. Ainsi, une modification de la décision d'exécution européenne relative aux mesures de lutte a été votée jeudi 19 octobre par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

La « stratégie bioéconomie pour la France » et les nombreuses études sur le sujet font ressortir que le développement de filières locales de matériaux biosourcés est l'une des composantes essentielles de l'avenir des territoires et de notre pays. Ces filières présentent également l'intérêt de pouvoir se mettre en place aux différentes échelles territoriales en s'appuyant sur des TPE et PME travaillant dans le cadre de démarches d'écologie industrielle et territoriale, voire de circuits courts. Par ailleurs, ces caractéristiques permettent aux collectivités locales d'agir directement sur les dynamiques de ces filières, au bénéfice de leur développement socio-économique.

emblématique de l'ensemble de la filière, depuis la culture du chanvre jusqu'à la production de matériaux isolants pour la construction. Aujourd'hui, la réussite significative de ces filières se heurte toutefois à trois obstacles majeurs d'abord, des cadres normatifs et réglementaires peu adaptés à leurs spécificités et à leurs dimensions ; ensuite, la grande difficulté à financer et à amortir les coûts de développement

le développement significatif des filières locales biosourcées ne pourra se faire sans un soutien fort des pouvoirs publics. Monsieur le ministre, quelles dispositions réglementaires, fiscales, financières d'accompagnement de l'innovation et de politiques d'achats publics

vous appelez mon attention sur la « stratégie bioéconomie pour la France » et m'interrogez plus spécifiquement sur les dispositions prévues par le Gouvernement pour favoriser le déploiement des matériaux biosourcés, notamment dans la construction. Je vous confirme que le développement de la bioéconomie est l'une des priorités de la stratégie gouvernementale. Un atelier y a d'ailleurs été consacré dans le cadre des états généraux de l'alimentation, que j'ai l'honneur de piloter, de piloter, dont le premier chantier est axé sur la création et la répartition de la valeur. Les présidents de cet atelier soulignent dans leurs conclusions l'importance de la stratégie nationale bioéconomie et la nécessité de faire aboutir le plan d'action qui en découle. Développer la filière biosourcée passe d'abord par une valorisation accrue de la biomasse, ce qui offre de nouveaux débouchés aux agriculteurs et aux forestiers, crée des emplois locaux de transformation de cette biomasse en matériaux et contribue à la transition vers une économie décarbonée. La bioéconomie est aussi un vecteur important de complément de revenu pour nos agriculteurs et nos forestiers, donc de meilleure valorisation de la biomasse française. Afin de favoriser la pénétration des matériaux biosourcés sur les marchés, plusieurs actions peuvent être mises en oeuvre : prendre en compte le caractère biosourcé dans les marchés publics, communiquer auprès du grand public, du grand public, sensibiliser le consommateur en créant par exemple un label ou un logo dédié qui lui permettrait de prendre en compte le caractère renouvelable des matières premières dont sont constitués les produits.

Il s'agit là d'un enjeu fort de la gestion du foncier : la préservation de nos terres agricoles est un objectif majeur, qui mérite de faire l'objet d'un traitement approfondi. Mesurant l'importance du rôle des SAFER, j'ai souhaité vous interpeller, monsieur le ministre, sur ce qui est, à mes yeux, un problème central. Il faut bien appréhender les difficultés

le modèle de financement des établissements publics fonciers est assis sur la contribution de l'ensemble du territoire de compétence de l'EPF. Par ailleurs, le désengagement financier de l'État depuis 2006, qui va une nouvelle fois s'accroître en 2018, limite encore plus les capacités d'action des SAFER,

pour le développement de l'agriculture en France, le renouvellement des générations, la régulation et la maîtrise du marché foncier rural, le développement local et la préservation de l'environnement. Le rôle des SAFER en qualité d'opérateurs fonciers a d'ailleurs été réaffirmé aout 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a notamment renforcé leurs modalités d'intervention- extension du droit de préemption des SAFER à l'usufruit et à la nue-propriété de biens ruraux et à l'intégralité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, à certaines certaines donations faites au profit d'une personne extérieure à la famille du donataire. Outre les rémunérations perçues sur les opérations qu'elles réalisent, les SAFER bénéficiaient d'une subvention publique. Ce financement, dont la suppression a été décidée par le Gouvernement en 2016, a fait l'objet de diverses mesures compensatoires d'ordre financier et fiscal. Par ailleurs, un financement est maintenu depuis 2017 pour les SAFER qui présentent des difficultés d'accès au marché foncier agricole, en l'occurrence les SAFER de Corse, de Guadeloupe, Martinique et de la Réunion. À ce jour, il n'est pas envisagé de rétablir une logique de financement public des SAFER. En revanche, une réflexion globale sur l'ensemble des outils de régulation devrait intervenir en 2018. Comme vous le savez, une mission parlementaire sur le foncier est prévue et sera conduite par le député Potier. Ce sera également l'occasion de réfléchir au positionnement des SAFER, à leur statut actuel- je rappelle que ce sont

En effet, en prenant la décision de supprimer l'aide au maintien pour les agriculteurs bio en 2018, le Gouvernement envoie un signal négatif à l'ensemble de la filière, même si les aides à la conversion progressent. Pour justifier votre choix, vous avez évoqué le nécessaire financement du bio par le marché. Je pourrais partager cette approche si le marché était à maturité, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui.

Ce montant doit être réparti entre les aides à l'agriculture de montagne, l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, l'ICHN, les mesures agroenvironnementales, l'assurance récolte et l'agriculture biologique. Sur ce transfert, Régions de France estime nécessaire le fléchage de 180 millions d'euros vers le financement de l'aide au maintien des Nous serons loin du compte, et les régions devront assumer une prise en charge complémentaire. À titre d'exemple, pour la région Pays de la Loire, cela représentera 675 000 euros. Le Gouvernement met ainsi les régions en difficulté et prend le risque de créer des déséquilibres territoriaux préjudiciables aux filières et aux producteurs. Alors que nous prônons la mise en place d'une véritable économie circulaire, de circuits courts, de productions locales de qualité, de bio-économie, alors que nous fixons des objectifs ambitieux pour le bio, notamment en matière de restauration scolaire, alors que les importations de produits bio sont en forte hausse, votre message trouble tous les acteurs engagés.

en croissance de 20 % par rapport à 2015, et la progression se poursuit au cours du premier semestre de 2017. Au 30 juin 2017, plus de 51 000 opérateurs étaient engagés dans dont plus de 35 000 exploitations et 16 000 transformateurs, distributeurs et importateurs. Les surfaces cultivées en agriculture biologique étaient estimées à 1,77 million d'hectares au 30 juin 2017, hausse de 15 % par rapport à la fin de l'année 2016. Pour accompagner cette transformation des modèles de production, l'État a pris l'engagement de réserver dans le Grand Plan d'investissement 5 milliards d'euros pour les filières agricoles. Bien sûr, cela concernera pour partie les filières biologiques, en fonction des

si, et comment, elles souhaitent accompagner les exploitations déjà converties. Monsieur le sénateur, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, j'ai demandé la conclusion

dans les travaux qui sont conduits dans chaque filière. Les crédits ont triplé pendant la période de programmation des fonds européens 2014-2020 par rapport à la période 2007-2013. Le soutien aux producteurs biologiques passe également de l'agriculture biologique, qui sera prolongé et significativement augmenté. Les producteurs biologiques bénéficient également de l'ensemble des aides accordées à l'agriculture au titre de la PAC. Enfin, et c'est essentiel, les prix payés aux producteurs sont tout à fait convenables dans les filières biologiques. Prix Prix payés aux producteurs, aides publiques, crédit d'impôt, perspectives de croissance : les filières biologiques sont très largement soutenues, et c'est bien normal pour des productions qui sont plébiscitées par nos concitoyens. Monsieur le sénateur, le développement du bio est l'une

du ministre de la cohésion des territoires. Ma question porte sur un enjeu de sécurité majeur dans le secteur de la construction : la certification des armatures du béton. Le béton armé est aujourd'hui le matériau de construction le plus utilisé en France. L'incorporation d'armatures est indispensable

peut gravement mettre en péril la solidité structurelle d'un ouvrage. Une série d'accidents récents, survenus notamment dans mon département, rappelle l'urgence de renforcer le contrôle de la qualité de la fabrication et de la pose de ces armatures. La France est semble-t-il en retard sur ce plan, alors que d'autres pays européens, comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique, ont déjà introduit une certification obligatoire pour les entreprises fabriquant ou mettant en oeuvre ces armatures. Les professionnels de la construction ne comprennent pas le retard pris dans la réglementation française et s'en inquiètent. La sécurité des bâtiments doit être une priorité si l'on souhaite éviter de nouveaux drames humains.

Seules 50 % des entreprises du secteur sont aujourd'hui titulaires de cette certification. À ce stade, le seul moyen d'assurer la sécurité des ouvrages serait de rendre obligatoire la certification

Je souhaiterais appeler l'attention sur l'application trop stricte de la réglementation concernant les préenseignes au bord des voies de circulation, dont l'installation est limitée par l'arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d'harmonisation des préenseignes dérogatoires. La mise en oeuvre de ce dispositif quelques difficultés, car la dérogation n'est accordée que dans des conditions restreintes, à savoir uniquement pour la vente de produits du terroir, les activités culturelles, les monuments historiques classés ouverts à la visite et les opérations et manifestations exceptionnelles, à titre temporaire. Or cette restriction de l'autorisation des préenseignes hors agglomération a des effets directs sur l'activité de petites entreprises, comme les restaurants et les hôtels, en particulier dans les territoires ruraux. Elle prive des professionnels d'une signalétique directionnelle indispensable au maintien de leur activité, la seule clientèle locale n'étant pas suffisante. Le chiffre d'affaires dépend en partie de la clientèle détournée des grands axes de circulation grâce à la préenseigne installée avant la bifurcation permettant d'accéder

Aussi ces entrepreneurs souhaiteraient-ils trouver, avec les services de l'État, une solution mieux adaptée à leur situation, afin que leur disparition de nos territoires Ma question, monsieur le ministre, est la suivante : peut-on alléger cette réglementation, qui constitue une nouvelle menace pour l'emploi ? Il y va de la survie de l'activité économique dans nos territoires, surtout dans les territoires ruraux.

en substitution aux préenseignes devenues illégales. Cette signalisation doit obligatoirement faire l'objet d'un schéma départemental ou communal,

Seul Orange tient plus ou moins ses engagements, alors que SFR annonce au contraire 100 % de couverture en 2025, sans aucune concertation, et que Bouygues et Free sont très en retrait en termes d'investissements.

territoires. Monsieur le sénateur, vous avez compris que le numérique est une grande priorité du Gouvernement, compte tenu de la situation que nous avons trouvée

et des villes moyennes, des bourgs-centres, des communes rurales qui se sentent oubliés alors qu'ils représentent près de 90 % du territoire français. Les ambitions affirmées en faveur des métropoles ne peuvent avoir pour conséquence de pénaliser l'immense majorité du pays. Afin de préserver un certain équilibre de notre territoire, il est donc primordial que les communes rurales puissent se développer et accueillir de nouvelles populations. Elles jouent un rôle majeur dans l'installation des jeunes,

perspective, la rénovation de l'habitat existant et la construction de manière responsable de nouveaux logements sont indispensables. S'il est admis que seule une fiscalité attractive pour les ventes de terrains incite à la construction, pourquoi réserver le bénéfice de ces mesures aux seules métropoles ? et de prévoir la réalisation d'un rapport d'évaluation des zones géographiques éligibles au PTZ devant permettre d'améliorer la pertinence des critères retenus. Toutefois, ces mesures ne seront pas suffisantes pour parvenir à un véritable équilibre territorial entre l'urbain et le rural. Comment comptez-vous, monsieur le ministre, soutenir les communes rurales et les villes moyennes qui souhaitent développer leur offre de logements ? Envisagez-vous de revoir les mécanismes de défiscalisation afin de permettre l'investissement les secteurs ruraux ?

rappelé la situation parfois difficile de certaines villes moyennes et de certains territoires ruraux. Que ne s'en est-on ému plus tôt ?

Certes, la situation des communes rurales et des bourgs-centres n'est pas nouvelle. Pour autant, je pense que nous devons tous agir pour l'améliorer et préserver la capacité

Connaissant bien la situation des territoires fragiles, dans les quartiers prioritaires mais aussi dans les départements ruraux, dont je suis issu, je sais que nous devons pouvoir nous appuyer sur un certain nombre de procédures adaptées.

sur la valeur ajoutée dans le cadre des opérations de transport scolaire. En effet, l'administration semble estimer que, si la somme des participations financières perçues par le conseil régional auprès des familles des élèves est supérieure à 10 % du coût de revient annuel des prestations relatives à l'ensemble des contrats de transport scolaire, cette contribution constitue « une relation directe entre la somme acquittée par les familles et la prestation de transport », d'où la possibilité de récupérer la TVA après assujettissement. L'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public, l'ANATEEP, que je préside, s'inquiète fortement des conséquences d'une telle règle pratique. deux tiers des départements ne laissent à la charge des parents d'élèves que de 0 % à 10 % du coût total annuel par élève transporté, soit quelques dizaines d'euros sur un coût total annuel de 1 000 euros. cette simple mesure aura donc pour conséquence inéluctable une remise en cause généralisée de la « gratuité » assurée jusque-là, les régions étant incitées à éviter la « double peine », à savoir financer la part familiale tout en renonçant à récupérer la TVA. J'ajoute que, pour des familles souvent en situation difficile, devoir payer 100 euros ou plus annuellement par enfant transporté constitue une dépense élevée. Compte tenu de la réalité sociale du service public de transport scolaire, qui concerne chaque jour 4 millions d'élèves, je vous demande de reconsidérer ce seuil de 10 %, si préjudiciable indirectement aux familles. Celui-ci apparaît excessif si l'on se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour ce type de services, puisqu'elle a estimé récemment qu'une part familiale de seulement 3 % entraînait la reconnaissance du caractère gratuit du service public de transport d'élèves. La parole est à M. le secrétaire

la fourniture, par une région, de prestations de transport de personnes à titre onéreux doit être soumise à la TVA lorsqu'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Pour cela, le bénéficiaire de la prestation doit en retirer un avantage individuel et le niveau de cet avantage doit être en relation avec le prix payé par la personne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne que vous évoquez ne fixe pas de seuil de contribution en pourcentage du coût des prestations au-delà duquel une prestation devrait être regardée comme entrant dans le champ d'application de la TVA. Par le passé, la Cour de justice la qualité d'assujetti à une personne publique dont les revenus tirés d'une activité d'assistance juridique ne couvraient que 8 % des coûts engagés. C'est pourquoi, en l'état de la jurisprudence, il a été considéré, à titre de règle pratique, que lorsque la somme des participations financières perçues par un conseil régional auprès de familles d'élèves était supérieure à 10 % du coût de revient annuel des prestations relatives à l'ensemble des contrats de transports scolaires, cette participation était de nature à caractériser l'existence d'une relation directe entre la somme acquittée par les familles et la prestation de transport fournie par ce conseil régional. Par ailleurs, je tiens à rappeler que lorsqu'un conseil régional accomplit, dans le cadre de son activité de transports scolaires, une opération de transport à titre gratuit, cette prestation est d'ores et déjà placée hors du champ d'application de la TVA, puisque le caractère onéreux, par définition, fait défaut. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de reconsidérer la décision, dans la mesure où la fixation d'un seuil qui serait inférieur à 10 % du coût de revient de la prestation de transport exposerait la France à un risque de contentieux communautaire important. Les travaux menés sur ce sujet par la direction des affaires juridiques de mon ministère

La Seine-Saint-Denis n'échappe pas à cette cure d'amaigrissement. Des fermetures avaient été annoncées l'an dernier, mais, devant la mobilisation des élus et de la population, des promesses de sauvegarde avaient été faites par le ministre des finances de l'époque. Or, en juillet dernier, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis nous a informés que les trésoreries d'Aubervilliers et de La Courneuve fermeraient leurs portes le 1 janvier 2018 pour se regrouper sur un seul et même site, à savoir celui d'Aubervilliers. La trésorerie de Bagnolet, à la fois trésorerie municipale et centre des impôts, serait, quant à elle, déplacée à Montreuil. D'autres sites, à terme, seraient également concernés. Ces fermetures sont dictées par une logique économique qui vise à supprimer la moitié des trésoreries d'ici à cinq ans pour, nous dit-on, alléger la facture de l'État. Cette logique n'est pas la nôtre. En Seine-Saint-Denis, nos villes cumulent déjà de nombreuses difficultés en matière d'accès aux services publics, comme La Poste ou les hôpitaux, pour ne citer que ces exemples. Les Séquano-Dyonisiens ont droit, au même titre que l'ensemble de la population, à un service public de proximité, fondé sur que les services dématérialisés ne peuvent pas remplacer. Demain, les Courneuviens devront se déplacer à Aubervilliers, où la trésorerie est surchargée, pour payer la cantine de leurs enfants ou acheter des timbres fiscaux. Cela vaudra également pour les usagers de Tremblay-en-France, de Stains ou encore d'Épinay-sur-Seine. Dans tous les cas de figure, les conditions d'accueil de ces usagers aussi bien que les conditions de travail des agents s'en trouveront fortement dégradées. Je me permets donc, ce matin, de relayer la colère qui s'exprime dans mon département par la voix des élus et des populations, qui refusent la fermeture et la fusion de ces services publics de proximité, et vous demande, monsieur le secrétaire

de l'économie et des finances. Madame la sénatrice, vous le savez, une action publique et un service public modernes et efficaces adaptent leurs implantations physiques aux évolutions démographiques, aux nouvelles technologies, aux nouveaux usages et à la nouvelle pratique des services publics de nos concitoyens. À l'évidence, cette pratique a évolué, au regard notamment du développement du numérique. Dans un monde où plus d'un contribuable sur deux déclare ses revenus en ligne, la qualité du service public ne se mesure pas strictement- cela ne veut pas dire que cet élément n'est pas important -à la seule présence physique sur le territoire.

Les populations les plus fragiles ou les plus éloignées de ces moyens de communication font l'objet d'un accompagnement particulier : des solutions innovantes peuvent être trouvées, comme la mise en place de permanences ambulantes sur des parties de territoire qui seraient mal couvertes. La DGFiP a en outre considérablement développé son offre de services à distance avec des permanences téléphoniques assurées selon des plages horaires étendues. La Seine-Saint-Denis est l'un des premiers départements couverts par un centre de contact, dispositif qui a pour objectif de faciliter la gestion à distance de la relation avec les usagers. Les deux projets de regroupement de trésoreries sont des reports d'opérations présentées en 2016, avec une date d'effet initialement prévue en 2017. La maturité insuffisante des projets a dicté ce report, afin que ces deux opérations puissent se dérouler dans les meilleures conditions à la fois pour les usagers et pour les agents. S'agissant de la trésorerie de La Courneuve municipale, son regroupement avec la trésorerie d'Aubervilliers s'inscrit dans une logique de rationalisation du réseau du secteur public local départemental. Compte tenu des distances réduites entre les communes de La Courneuve et d'Aubervilliers, l'incidence pour les usagers nous paraît limitée. Le regroupement de l'activité « secteur local » de la trésorerie de Bagnolet avec la trésorerie spécialisée de Montreuil municipale permettra de renforcer la qualité des prestations de conseil apportées par le comptable public. public. Le passage en comptabilité commerciale de l'office public de l'habitat de la commune a notamment eu pour conséquence une baisse importante d'activité de cette trésorerie. Par ailleurs, le regroupement au sein du service des impôts des particuliers de Montreuil et du recouvrement de l'impôt permettra aux usagers concernés de bénéficier d'un interlocuteur unique pour leurs questions portant sur l'assiette et le recouvrement de leurs impôts. Un site a déjà été identifié. Enfin, comme pour l'opération précédente, compte tenu des distances réduites entre les communes de Bagnolet et de Montreuil, l'incidence pour les usagers nous paraît également limitée. La direction départementale des finances publiques a néanmoins manifesté son accord

mais les faits sont têtus. Il y aura des fermetures de trésoreries en Seine-Saint-Denis ; cela va toucher des populations défavorisées, mais aussi les agents de ces structures, qui créent souvent du lien avec les populations et sont très à l'écoute des situations parfois difficiles que vivent des hommes et des femmes de ce département.

des services du ministère de la culture, selon sa valeur et son ancienneté. Cette réglementation s'applique aux professionnels comme aux particuliers, et c'est bien normal. L'exportateur doit alors remplir un formulaire, qui diffère suivant que le pays de destination

Le premier est de permettre la protection des oeuvres les plus importantes, que l'État peut qualifier de trésors nationaux. Le second est de contribuer à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, qui a pris une ampleur particulièrement préoccupante, depuis quelques années, dans la zone moyen-orientale. Depuis l'ouverture du marché unique européen en 1993, l'exportation des biens culturels hors du territoire douanier national est subordonnée à une double réglementation : une réglementation nationale et une réglementation communautaire. La France a fait le choix de calquer le champ d'application national sur le champ d'application européen : les autorisations sont exigibles pour les mêmes biens répartis entre quinze catégories, assorties de seuils de valeur et d'ancienneté, tout cela étant cumulatif. Cette préoccupation concernant les seuils est prise en compte par le Gouvernement, qui doit cependant veiller à leur proportionnalité et à leur équilibre en fonction de deux enjeux : garantir un bon niveau de protection du patrimoine, ce qui peut parfois des seuils bas pour certaines catégories, et ne pas faire peser des contraintes trop lourdes sur les opérateurs, pour ne pas entraver le développement du marché français de l'art. les délais, des retards ont effectivement été constatés. Il convient d'avoir conscience que les vérifications nécessaires préalables à la délivrance de tels certificats

Quant au relèvement des seuils pour certaines catégories nationales, sachant que les catégories communautaires restent inchangées, le Gouvernement a décidé de relancer, en l'actualisant, le travail qui a été réalisé il y a quelques années en vue de modifier l'annexe

est obligatoire pour tous les étudiants scolarisés dans un établissement d'enseignement supérieur âgés de seize à vingt-huit ans et ne bénéficiant pas du régime spécial d'un membre de leur famille.

Ainsi, certains étudiants ont le privilège de rester plus longtemps que d'autres affiliés au régime de leurs parents. Des régimes spéciaux peuvent en effet dispenser d'affiliation au régime étudiant jusqu'à l'âge Ce système de gestion du RSSE fait constamment l'objet de critiques au regard des inégalités qu'il crée selon les catégories d'étudiants, mais également des difficultés de gestion récurrentes de ses structures. Alors que la réforme de ce régime d'assurance maladie des étudiants annoncée par le Président de la République au cours de sa campagne semble plus que jamais d'actualité, notamment à la suite des annonces relatives au plan Étudiants du Gouvernement, je souhaiterais connaître, madame la secrétaire d'État, les modalités de sa mise en oeuvre

avec le Président de la République. À titre liminaire, il me paraît utile d'émettre une réserve d'ordre sémantique sur la dénomination « régime de sécurité sociale étudiant », qui est généralement utilisée pour désigner le dispositif d'affiliation des étudiants et de service des prestations qui leur sont dues, en ce qu'elle est juridiquement fragile. En effet, les étudiants sont affiliés par la loi au régime général de la sécurité sociale et la délégation de gestion dont bénéficient les mutuelles étudiantes n'est pas, en soi, constitutive d'un régime de base. S'agissant de la délégation de gestion accordée aux mutuelles d'étudiants, le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, dont le Parlement sera prochainement saisi, prévoit de mettre fin à ce dispositif spécifique dans un délai de deux années au plus tard et de replacer en conséquence les étudiants dans le droit commun, en cohérence avec la logique de la protection universelle maladie. L'objectif de cette réforme est de simplifier les procédures d'affiliation des étudiants, qui sont actuellement complexes et qui leur imposent, dans la majorité des cas, de changer d'organisme gestionnaire et de carte Vitale lors de leur inscription dans l'enseignement supérieur. Cette réforme doit permettre aux nouveaux étudiants d'être, à l'avenir, des assurés autonomes affiliés au régime de protection sociale de leurs parents et de bénéficier ainsi de la même qualité de service que les autres assurés. Tel n'était pas le cas jusqu'ici, comme l'ont établi de nombreux rapports. À compter de la rentrée 2018, les nouveaux entrants dans l'enseignement supérieur resteront ainsi rattachés pour le remboursement de la part de base de leurs frais de santé aux organismes qui géraient auparavant leur couverture maladie. Les autres étudiants, qui étaient précédemment rattachés à une mutuelle d'étudiants pour leur couverture de base, resteront rattachés à la même mutuelle pendant l'année universitaire 2018-2019. Au 1 septembre 2019 au plus tard, s'ils sont toujours étudiants, ils seront rattachés aux caisses du régime général. Les mêmes règles devraient être retenues pour les étudiants dont les parents sont affiliés à un régime spécial. En cohérence avec ces évolutions, la cotisation de 217 euros qui est actuellement demandée aux étudiants sera supprimée dès la rentrée 2018 et remplacée par une contribution unique « vie étudiante ». Cette mesure se traduira,, pour l'ensemble de la population étudiante, par un gain de pouvoir d'achat global de 100 millions d'euros.

du Léman, centre hospitalier situé à Thonon-les-Bains, dans le Chablais, en Haute-Savoie, un département que vous connaissez bien, madame la secrétaire d'État. Cet ensemble hospitalier de 730 lits constitue la seule offre de soins du bassin de vie chablaisien, qui compte 143 000 habitants. Ce territoire, fortement touristique, marqué par une dynamique démographique soutenue, présente une facette urbaine, autour du Léman, et une autre montagneuse, avec les stations de sports d'hiver. Le maintien des activités de soins de proximité prodiguées par les Hôpitaux du Léman est donc essentiel au regard des besoins de ce territoire. Or, depuis plusieurs mois,

de santé. Aujourd'hui, cet établissement n'a plus la capacité financière de se restructurer, de se moderniser et de maintenir dans un état décent ses équipements. Les photographies que j'ai adressées à Mme la ministre en témoignent. Cette incapacité de projection contribue largement à une hémorragie de son personnel avec, pour corollaire évident, une aggravation de ses pertes financières.

Il craint une disparition programmée de son outil de travail. C'est pourquoi je souhaite connaître vos propositions pour accompagner les Hôpitaux du Léman dans une dynamique positive lui permettant d'offrir rapidement de meilleures conditions d'accueil et de travail et d'assurer ainsi sa pérennité, alors que le M. le Premier ministre s'est engagé,

à une situation financière dégradée, s'expliquant pour partie par l'impact de la réforme du régime des transfrontaliers et la baisse d'activité, dans un environnement concurrentiel, ainsi que par un défaut de performance global, un plan de redressement est en cours d'élaboration.

Les aides octroyées en 2017 ont notamment permis de commencer certains travaux d'aménagement du site principal sis à Thonon-les-Bains, qui nécessiterait plus globalement une remise aux normes, avec une adaptation de l'établissement aux nouvelles pratiques médicales, notamment ambulatoires, dans un contexte de forte évolution démographique locale. À ce titre, un projet de reconstruction du bâtiment d'hébergement principal avait déjà été élaboré, pour un montant estimé à 80 millions d'euros, permettant ainsi de parachever la modernisation engagée en 2012 avec la mise en service du nouveau bâtiment de médecine. La perspective de cet investissement reste d'actualité, et un projet soutenable accompagnant le plan de redressement doit aujourd'hui être travaillé et construit en différentes phases, en tenant compte des priorités les plus immédiates, mais également du projet territorial du groupement hospitalier de territoire élaboré par le centre hospitalier Alpes-Léman. Ces objectifs figureront dans la feuille de route du prochain chef d'établissement, actuellement en cours de recrutement. Celui-ci devra aussi renouer des liens opérationnels avec la communauté médicale d'établissement et, plus globalement, la communauté hospitalière, afin d'engager un portage institutionnel des différents projets. La recherche de solutions pérennes passera aussi par la constitution d'équipes médicales de territoire dans le cadre du groupement hospitalier de territoire. Une procédure adaptée a déjà été mise en place par les

vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, les Hôpitaux du Léman peuvent s'appuyer sur un certain nombre d'atouts pour enclencher une dynamique positive : un territoire à forte croissance démographique,

Madame la ministre, ma question concerne la problématique des déserts médicaux. En effet, malgré les mesures mises en oeuvre par les gouvernements successifs, l'accès aux soins demeure difficile pour un grand nombre de nos concitoyens, particulièrement en milieu rural. Certains spécialistes font cruellement défaut. Par exemple, dans mon département, le Cantal, les délais pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue dépassent une année. Il ne reste plus que deux urologues dans le département. Les pédiatres, les gynécologues, les pneumologues se font rares, même à l'hôpital public. Nombre de nos concitoyens sont contraints de tenter d'obtenir des rendez-vous à Clermont-Ferrand, à plus de deux heures et demie de route de chez eux. Quelles mesures peut-on envisager pour pallier ces difficultés ? La situation de la médecine générale est également très préoccupante dans nos zones de montagnes. Beaucoup de médecins partent à la retraite et leurs cabinets médicaux ne sont souvent pas repris. Des maisons de santé ont certes été mises en service, mais encore faut-il réussir à trouver des médecins pour s'y installer. Or cela reste un exercice très difficile. Un élément qui semble freiner considérablement l'installation de jeunes généralistes en zone de montagne est le problème des astreintes les territoires à couvrir sont très vastes en raison de la faible densité de population et les conditions climatiques peuvent être très difficiles, voire hostiles, en particulier la nuit au coeur de l'hiver. Comment lever ce frein à l'installation ? Ne serait-il pas possible de renforcer et d'impliquer plus fortement encore les services des urgences de nos hôpitaux de proximité ?

Répondre aux besoins légitimes des Français en matière de santé est un impératif, comme vous l'avez souligné. Nombre de nos concitoyens n'y ont toujours pas accès dans un délai raisonnable. Il n'existe pas de solution unique ou uniforme. Beaucoup de choses ont été faites, mais il nous faut aller plus loin. Pour lutter contre les déserts médicaux, il est nécessaire en effet de disposer d'un panel de solutions adaptées aux territoires. Les maisons de santé pluridisciplinaires sont une solution et, conformément à l'engagement du Président de la République, nous en doublerons le nombre. Mais ce n'est pas la seule Il nous faut accélérer le déploiement de la télémédecine et de la santé numérique en général. Il faut aussi mettre en valeur les innovations locales, qui sont nombreuses. Agnès Buzyn souhaite également développer les pratiques avancées des professionnels de santé, notamment paramédicaux. Le Gouvernement souhaite encourager la possibilité que des médecins détachés depuis l'hôpital tiennent des consultations dans des zones sous-dotées. De même, il faut explorer la possibilité que des praticiens libéraux puissent assurer une consultation temporaire dans ces mêmes zones sans forcément s'y installer. Cela ne peut se faire sans une coordination de tous les acteurs de terrain, professionnels de santé, agences régionales de santé et collectivités locales. Il nous faut des solutions concrètes qui apportent des réponses en termes de pertinence des soins et de qualité de prise en charge des usagers. Agnès Buzyn souhaite donner à l'ensemble des acteurs tous les moyens afin qu'ils puissent organiser ou réorganiser les soins sur l'ensemble de nos territoires. Tout ce travail prendra du temps, et plusieurs mesures s'inscriront dans le temps long. Mais des solutions à court terme sont également proposées, car il nous faut répondre à l'urgence. C'est le but du plan territorial d'accès aux soins présenté le 13 octobre dernier. Un comité de suivi vient compléter ce plan afin de garantir son succès.

Par manque de courage politique, par méconnaissance de la réalité de nos territoires, ce gouvernement, qui se veut pourtant le chantre d'un nouveau monde, a décidé de poursuivre, en matière de lutte contre les déserts médicaux, la vieille politique, celle qui ne repose que sur les incitations et qui a démontré depuis vingt-cinq ans son inefficacité. Comment ne pas être déçu de ces choix, alors que l'accès aux soins se dégrade d'année en année ? Selon une étude récente, 148 cantons ne comptent plus aucun médecin généraliste, alors que ce chiffre était de 91 en 2010. Le département de l'Eure, dont je suis élu, compte 1,7 médecin pour 1 000 habitants, contre 7,5 à Paris, soit un rapport de un à

les délais étant beaucoup plus longs dans de très nombreux cas. Selon un sondage, cette situation conduit à ce que 70 % des Français renoncent à se faire soigner, compte tenu des délais auxquels ils sont confrontés. Devant ce constat, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable demande la mise en place d'un conventionnement sélectif, selon le principe « une installation pour un départ » dans les zones surdotées. Ce système a été mis en place pour d'autres professions de santé- infirmiers, sages-femmes, orthophonistes et chirurgiens-dentistes -et a prouvé son efficacité. Aujourd'hui, son extension aux médecins est de plus en plus souhaitée par les associations d'élus et les parlementaires. Des amendements au PLFSS allant en ce sens ont été signés par 110 sénateurs. Je vous le dis

Comptez-vous faire un bilan des mesures qui ont été annoncées et, si oui, à quelle échéance ? Dans l'hypothèse où les craintes que je viens d'exprimer se confirmeraient, envisagez-vous d'entendre nos propositions en matière de régulation de l'installation, mais aussi de formation des futurs médecins- il y a beaucoup à dire en la matière -, ou comptez-vous rester dans le déni de la réalité, jusqu'à ce qu'un drame sanitaire vous oblige à agir enfin ?

présenté au côté du Premier ministre, le 13 octobre dernier, un plan territorial d'accès aux soins ambitieux et pragmatique. Ce plan s'appuie sur le terrain, sur les remontées des professionnels de santé, des collectivités territoriales et des usagers. Pour remédier aux difficultés que rencontrent nos concitoyens en matière d'accès aux soins, il n'y a pas de réponse miracle, mais un panel de solutions. Ce plan représente un vrai changement de paradigme. L'accès aux soins repose non pas sur l'installation d'un médecin, mais sur l'organisation coordonnée entre tous les professionnels de santé du territoire. Ces solutions doivent être trouvées au niveau local, dans chaque territoire, par les acteurs eux-mêmes : il faut donc leur donner le maximum de liberté d'organisation. Le plan d'accès territorial aux soins ne s'appuie pas sur la coercition, car elle est contre-productive.

Le plan a pour objectif d'augmenter le temps consacré aux soins des professionnels de santé en levant les freins réglementaires qui empêchent les acteurs de terrain d'innover et de répondre aux besoins de la population, et surtout de répondre de manière rapide à la problématique de l'accès aux soins. Ce plan Ce plan généralisera la téléconsultation et la télé-expertise, en permettant aux professionnels les pratiquant d'être rémunérés et en équipant tous les EHPAD et toutes les zones sous-denses d'ici à 2020. Il faut accompagner la mise en place de la télémédecine. Ce plan favorisera aussi la coopération entre professionnels de santé, en doublant le nombre des maisons de santé pluriprofessionnelles en cinq ans grâce à un programme d'investissement de 400 millions d'euros dans le cadre du Grand Plan d'investissement. Agnès Buzyn souhaite aussi développer les consultations avancées et créer des postes d'assistant partagé. Le cumul emploi-retraite pour les médecins installés est inscrit dans le PLFSS pour 2018. De nouvelles aides conventionnelles destinées à favoriser l'installation des médecins dans les zones sous-denses verront le jour : elles s'élèveront à 50 000 euros sur trois ans pour l'installation d'un médecin dans une souhaitons également valoriser les contrats conventionnels dans le cadre des zones sous-denses, dont le contrat de solidarité territoriale médecin, visant à inciter à la réalisation de consultations avancées dans les territoires qui en ont le plus besoin. Ce plan sera amené à évoluer en fonction des besoins de la population et des évolutions démographiques. Trois délégués ont été nommés pour intégrer le comité de suivi : M. Thomas Mesnier, député, Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, et Mme Sophie Augros,

pour répondre aux difficultés croissantes de recrutement dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Malgré les nombreuses initiatives qu'ils mettent en oeuvre, la situation des EHPAD devient intenable.

Les entreprises du secteur ont besoin de soutien, d'une part pour valoriser les métiers et les carrières qu'elles promeuvent, d'autre part pour professionnaliser l'accompagnement en gérontologie. Avec un potentiel d'environ 350 000 emplois à l'horizon 2030, le secteur du grand âge enregistre pourtant une pénurie de personnel soignant. Aussi je crois vraiment indispensable de lever les freins spécifiques au recrutement dans cette filière, en assurant une promotion coordonnée avec Pôle emploi, les régions, l'État et les acteurs du secteur. La création d'une véritable filière professionnelle des métiers du grand âge, avec un métier de soignant spécialisé, permettrait également une meilleure intégration de la gériatrie et de la gérontologie dans les cursus médicaux et paramédicaux. Madame la secrétaire d'État, alors que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus représentera plus d'un tiers de la population française en 2060, contre un quart aujourd'hui, et que l'augmentation la plus forte concernera les plus âgés-

Ils représentent 70 % des établissements dédiés à l'hébergement des personnes âgées, 53 % d'entre eux faisant partie du parc hospitalier public. Je tiens tout d'abord à saluer le travail réalisé au quotidien par les personnels dans les EHPAD. Chacun et chacune, à leur niveau- soignants, accompagnants, animateurs, personnes chargées de l'hôtellerie, de l'accueil ... -, participent à la prise en charge des personnes âgées au sein de notre société et leur donnent une place à part entière parmi nous.

à l'adaptation de la société au vieillissement met en oeuvre un plan des métiers de l'autonomie. Ce plan a pour objet de rendre les métiers du secteur plus attractifs et d'offrir aux salariés un véritable parcours professionnel. Les personnels des EHPAD participent au repérage de la maltraitance. Un programme national de contrôle préventif des établissements médico-sociaux au titre du repérage des risques de maltraitance est mis en oeuvre. Toutefois, nous entendons lui donner un souffle nouveau, avec la mise en place d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la maltraitance afin de renforcer la prévention. Un nouveau plan d'action sera arrêté au second semestre de 2018, après concertation et apport des réflexions du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Agnès Buzyn salue le rôle central joué par les personnels des EHPAD pour prévenir les cas de maltraitance au sein de leurs établissements. Pour répondre aux besoins de notre population et aux évolutions démographiques, le PLFSS pour 2018 prévoit 4 525 places supplémentaires d'hébergement permanent en EHPAD.

Enfin, les conditions de travail des personnels, et particulièrement des soignants, sont souvent difficiles. C'est pourquoi nous avons lancé une mission importante sur la qualité de vie au travail et la formation, afin de leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions leur mission au chevet de nos aînés. Vous pouvez compter sur notre vigilance.

Mon compagnon est parti précipitamment pour passer la nuit auprès du troupeau, en ayant l'intention de dormir dans la voiture, sachant qu'il est prévu moins de zéro degré cette nuit. « Suite à l'attaque que nous avons subie dimanche dernier, et la perte de 15 brebis sur notre troupeau de 150 têtes, nous ne pourrons pas supporter de pertes supplémentaires. Le troupeau est actuellement très stressé, nous craignons des avortements. Quelle profession peut accepter cette pression ? Nous sommes désemparés. « Nous sommes installés depuis trois ans ; nous avons investi toute notre énergie, nos convictions et nos finances dans notre projet d'élevage de brebis avec valorisation en vente directe des agneaux et de la laine, certifiés en agriculture biologique. Nous bénéficions d'un réel accueil et soutien local pour la remise en pâturage de collines et la vente de laine et de viande d'agneau. Nous avons mis en oeuvre, depuis notre installation, toutes les mesures de protection préconisées parcs électrifiés, chiens de protection, surveillances " pluriquotidiennes ". « Ce soir, je souhaite donc exprimer notre sentiment d'impuissance et de découragement face à la pression de prédation du loup, qui depuis quelques mois s'est nettement intensifiée dans le sud des Baronnies. « Ne sous-estimez pas l'urgence de la situation ! Nous avons besoin de réponses concrètes. le témoignage que j'ai reçu dernièrement à ma permanence. Je n'aurais pas pu poser plus clairement la problématique du loup dans nos territoires et exprimer de façon plus éloquente le désarroi des éleveurs. En Drôme, les chiffres les plus récents indiquent une augmentation de 31 % du nombre d'attaques et de bêtes tuées par rapport à 2016, après un doublement l'année précédente

par le ministère de l'environnement. Il indique que « dans tous les cas, l'état actuel de la population en France, en termes d'effectifs et de croissance, semble garantir la viabilité démographique ». Compte tenu de ces éléments scientifiques et du témoignage dont je viens de vous faire part, je souhaite, madame la secrétaire que vous me fassiez connaître les intentions du Gouvernement en matière de déclassement du statut du loup en vue d'une protection moins stricte et que vous m'indiquiez si vous envisagez d'entreprendre des démarches en ce sens au niveau européen.

Le loup est une espèce protégée, qui fait son retour en France depuis une vingtaine d'années. C'est une bonne nouvelle pour la biodiversité, qui est notre bien commun, mais c'est aussi un véritable défi pour les éleveurs qui font face à la prédation des loups. Dans ce contexte,

territoire et la protection des éleveurs. Nous comprenons la détresse et la souffrance de ceux qui sont confrontés aux conséquences des attaques sur leur troupeau. La méthode employée jusqu'ici n'était pas satisfaisante. Elle privilégiait le court terme, en autorisant l'abattage de quelques dizaines de loups chaque année de manière assez arbitraire.

concertation avec les acteurs. L'objectif est de sortir de la confrontation et de l'opposition binaire et de construire ensemble des solutions qui soient viables pour tous sur le long terme. Le Gouvernement a posé quelques principes pour cette concertation. Je le redis ici, ceux qui voudraient l'éradication de tous les loups et ceux qui nient la détresse des éleveurs doivent entendre raison. Par ailleurs, nous devons passer à une logique de protection et de défense des troupeaux pour aider les éleveurs, qui doivent pouvoir éviter les attaques, mais aussi se défendre. C'est pourquoi les tirs de défense et de défense renforcée doivent être privilégiés. C'est en quelque sorte de la légitime défense, mais cela ne peut se faire que si tout a été fait pour protéger les troupeaux avant. C'est aussi cela, la cohérence. Les études du ministère de l'agriculture montrent que les mesures de protection sont efficaces quand elles sont combinées présence du berger, chien de protection, parc de nuit, d'où la nécessité de les mettre en place y compris là où le loup n'est pas encore installé. La concertation se poursuit pour développer une panoplie d'outils obéissant à ces principes et le plan Loup du Gouvernement sera présenté au premier trimestre de 2018.

fondée sur le constat que certaines espèces protégées par la directive Habitats sont devenues des menaces pour d'autres espèces, en particulier pour les animaux d'élevage. Une brèche a donc été ouverte, et il serait important que la France s'y engouffre en sollicitant un changement de statut du loup

Je suis donc surprise que, à peine élu, le président Macron ait fait supprimer les aides de l'État au maintien de l'agriculture biologique. À la suite de ce revirement, un grand quotidien national a titré en ces termes : « Le Gouvernement pense notre lendemain avec les concepts d'hier ».

les services de l'État examinent actuellement un projet d'élevage industriel de 40 000 poulets en batterie sur 1 800 m, soit 21 poulets au mètre carré.

Peut-être me répondrez-vous qu'il convient de faire preuve de pragmatisme. Auquel cas je vous demanderai quelle est la frontière entre le pragmatisme et le renoncement ! En 1976, dans la comédie, le réalisateur Claude Zidi dénonçait déjà la nourriture industrielle et la malbouffe. Dans ce film, le critique gastronomique Duchemin, interprété par l'excellent Louis de Funès, faisait triompher la vérité face à l'infâme industriel Tricatel, qui cherchait à nous empoisonner pour faire du profit. ans plus tard, la fiction est malheureusement devenue réalité. Nous ingurgitons du faux fromage à base d'huile de palme et nous mangeons des manchons de poulet reconstitués à partir de déchets d'os recouverts de gel et de peinture alimentaire- j'ai personnellement assisté à leur fabrication Je doute que l'on prépare ce type de nourriture dans les cuisines de l'Élysée, mais, dans les salons ministériels, on doit malheureusement juger qu'elle est assez bonne pour nos enfants Plus qu'au ministre ou à son représentant, je m'adresse par votre intermédiaire, madame la secrétaire d'État, à Nicolas Hulot, au citoyen engagé qui s'est longtemps battu pour sensibiliser les Français à l'écologie et qui défendait un autre modèle de société.

transition écologique et solidaire. Madame la sénatrice, M. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, ne pouvant être présent, il m'a chargée de vous répondre. Votre question fait évidemment écho au vaste et important débat qui s'est ouvert dans le cadre des états généraux de l'alimentation. Ce que nous produisons et mangeons a des conséquences directes sur la planète et sur la vie de nos concitoyens. L'agriculture et l'alimentation sont créatrices de paysages, de richesses et de lien social. Dans le même temps, certaines évolutions des cinquante dernières années sont à l'origine d'impacts profondément négatifs sur l'environnement. Elles affectent ainsi les ressources et la biodiversité et participent au réchauffement climatique. Se posent aussi les questions de la pérennité de l'emploi agricole et de la rémunération des producteurs au regard de la récurrence des crises agricoles. De plus en plus conscients de ces enjeux, nos concitoyens sont demandeurs de produits alimentaires plus respectueux de l'environnement et souhaitent aussi la prise en compte du bien-être animal. Ils se préoccupent de l'origine des produits et appellent au renforcement des liens entre producteurs et consommateurs. Le ministre d'État attache la plus grande importance à ce que s'engage la transition écologique de l'agriculture. À ses côtés, nous ambitionnons que, à terme, la norme relève des principes de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Nombre d'agriculteurs sont aujourd'hui engagés ou prêts à s'engager dans cette voie. De multiples initiatives montrent que cette transition est possible, mais qu'elle doit être accompagnée. Les états généraux de l'alimentation, qui ont été lancés le 20 juillet dernier et sont pilotés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, impliqueront jusqu'à la fin de ce mois l'ensemble des parties prenantes. Ils devront établir un diagnostic partagé et proposer des solutions aux problèmes rencontrés par l'agriculture. Le 11 octobre dernier, le Président de la République a confirmé nos nouvelles orientations par une meilleure prise en compte des enjeux de qualité, de protection de l'environnement et du bien-être animal, elles doivent doter notre pays d'une stratégie visant à nous permettre de recouvrer notre souveraineté alimentaire. Le ministre d'État sera particulièrement vigilant à ce qu'émergent des propositions allant dans le sens d'une transformation en profondeur des modèles agricoles, en particulier pour les systèmes d'élevage. D'ores et déjà, différents chantiers progressent vers la transition écologique de l'agriculture. À ce titre, le Gouvernement s'engage à développer un plan de sortie des pesticides, qui constituent un autre grand sujet de préoccupation pour nos concitoyens.

Ces terres cultivables permettraient d'encourager en Île-de-France le développement des circuits courts et d'une production locale respectueuse de l'environnement, comme le propose notamment les auteurs du projet alternatif CARMA.

des temps de trajet, car les autoroutes A1 et A3, déjà surchargées, seront complètement saturées. L'autorité environnementale indique que le temps de trajet entre Paris

La mobilisation citoyenne grandit, à juste titre, contre EuropaCity et M. le ministre d'État Nicolas Hulot s'est lui-même prononcé contre la réalisation de ce projet -incompatible avec le plan Climat -, tout comme le commissaire enquêteur. Nous les rejoignons sur ce point nous ne souhaitons pas la réalisation de ce projet, qui véhicule un modèle de société contribuant à la mise à bas des objectifs de la France en matière de préservation

de la France en matière environnementale

Le projet d'extension urbaine de très grande ampleur que vous évoquez pose la question de la refondation de notre modèle d'aménagement commercial, pour le rendre plus respectueux de la préservation des espaces agricoles et naturels.

La desserte de ce complexe, malgré le projet de création d'une gare du futur Grand Paris Express, requerra de façon majoritaire le recours à la voiture. Cet aménagement contribuera donc à la congestion du trafic, déjà très dense dans ce secteur, à la dégradation de la qualité de l'air, mais aussi à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, l'implantation du projet est incompatible avec les objectifs de préservation des terres agricoles et de lutte contre l'artificialisation des sols inscrits notamment dans le schéma

Malgré plusieurs avis défavorables, le plan local d'urbanisme de la ville de Gonesse, révisé en octobre dernier, autorise l'ouverture à l'urbanisation du triangle de Gonesse. Le commissaire enquêteur a également rendu des conclusions défavorables, relayant des préoccupations de la population exprimées lors de la concertation. Pour toutes ces raisons, je ne peux que m'interroger sur la compatibilité du projet, dans son état actuel, avec les politiques de transition écologique et solidaire que Nicolas Hulot Nous avons néanmoins conscience que ce projet pourrait contribuer au développement économique régional, le triangle de Gonesse ayant été identifié comme un territoire stratégique pour le Grand Paris. Ce projet a été soutenu par le précédent gouvernement et continue d'être accompagné par un opérateur de l'État. Aussi semble-t-il nécessaire d'engager, sur ce dossier, un travail interministériel, en tenant compte des attentes des collectivités concernées,

Mon département, l'Aisne, est situé sur l'axe stratégique qui relie Paris à la Belgique, et constitue par conséquent une voie de passage très empruntée, que ce soit par route ou par rail. Malgré cet intérêt et cette forte fréquentation, ses infrastructures terrestres et ferroviaires ne bénéficient toujours pas des investissements nécessaires à leur pleine exploitation,

aux côtés de la SNCF, ou encore du maintien de la ligne de fret Fismes-La Ferté-Milon afin d'assurer la continuité de l'activité économique locale. Les collectivités territoriales ont mis la main à la poche, alors même que certaines ne sont plus concernées par cette compétence. L'État doit participer à cet effort,

Concernant la ligne ferrée Paris-Laon, comment compte-t-il préparer l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux de voyageurs, afin de concilier la prise de responsabilité croissante de la région et le maintien d'une infrastructure adéquate et performante ?

Nous souhaitons être pleinement rassurés à ce sujet, les usagers de la ligne Paris-Laon subissant d'ores et déjà des perturbations récurrentes -ponctualité déficiente, suppressions de trains, mauvais état de la ligne, etc.

Alors que cette semaine est dédiée aux maires de France, réunis en congrès à Paris, et que le président du conseil départemental de l'Aisne, Nicolas Fricoteaux, doit rencontrer le 28 novembre prochain votre collègue Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, pour évoquer les actions nécessaires au développement du territoire axonais, j'en appelle au Gouvernement pour qu'un oeil bienveillant

vous répondre. Je tiens à vous assurer de toute l'attention que porte l'État à la RN2. Le contrat de plan État-région 2015-2020 a d'ores et déjà inscrit la poursuite de l'aménagement de la RN2 dans l'Aisne, en particulier entre Paris et Laon. Plusieurs études et programmes d'amélioration d'itinéraires sont également en cours, en particulier à Silly-le-Long, sur la déviation de Soissons ou, au nord du département, sur la section de la RN2 comprise entre Laon et Avesnes-sur-Helpe. Concernant la ligne de TER Paris-Laon que vous avez évoquée, la régularité constatée sur cet axe, malgré une progression, reste encore insuffisante : cela tient largement à l'état vieillissant des infrastructures, qui nécessite la réalisation d'opérations lourdes de maintenance entraînant des ralentissements et un aménagement du plan de transport avec des substitutions routières, notamment le week-end.

Concernant l'ouverture à la concurrence des TER que vous avez mentionnée, la mission confiée par le Gouvernement à Jean-Cyril Spinetta vise précisément à en déterminer les conditions de réussite. Les conclusions de cette mission sont attendues pour le début de 2018.

Pour autant, l'ensemble des études déjà menées sur l'exploitation ferroviaire du CDG Express a montré la compatibilité de celle-ci avec ces différentes circulations, notamment celle du TER, qui pourra conserver ses horaires. La commission d'enquête publique l'a d'ailleurs confirmé. Soyez ainsi assuré, monsieur le sénateur, que, conformément aux priorités nationales qu'il s'est fixées, le Gouvernement entend bien apporter de réelles améliorations aux liaisons du quotidien, sur les réseaux tant ferroviaires que routiers.

les déplacements quotidiens des habitants de la métropole et le passage d'un trafic de transit français et européen. Les chiffres, qui ne cessent d'augmenter, sont éloquents et suffisent à traduire cette réalité, qui empoisonne le quotidien de milliers d'automobilistes : plus de 100 000 véhicules circulent chaque sur le pont d'Aquitaine, et plus de 140 000 sur la rocade est. La rocade bordelaise supporte des trafics moyens hors du commun, de l'ordre de 265 000 véhicules par jour. Chaque automobiliste communautaire doit consacrer 1 heure 20 à ses déplacements quotidiens. Il faut savoir que, de janvier à septembre, la circulation a augmenté de 2,5 % sur l'intrarocade rive droite et que, sur l'intrarocade Bordeaux-Nord, le trafic a progressé de plus de 3,3 %. En cinq ans, le trafic des poids lourds a crû de plus de 12 %. Une telle saturation du trafic se traduit d'ores et déjà par le gaspillage d'au moins 60 000 heures, perdues quotidiennement sur la rocade, et, au-delà, par des conséquences économiques et environnementales dont je chiffre le coût à près de 1 million d'euros par jour. Quotidiennement, le point noir routier de Bordeaux est cité sur toutes les radios. Plus de 3,5 millions de déplacements sont effectués quotidiennement à l'intérieur de l'agglomération bordelaise et les projections les plus sérieuses annoncent une progression effrayante, plus de 2 millions, du nombre de ces déplacements, ce qui fait craindre le pire. On aurait pu espérer que les travaux d'élargissement de la moitié sud de la rocade ouest, ainsi que les travaux

qui a été abandonné à cause des conclusions du Grenelle de l'environnement. Au moment où le président de la métropole bordelaise, Alain Juppé, pointe la nécessité urgente de réaliser une telle infrastructure,

que l'on peut désormais rejoindre Paris en deux heures, alors que l'on peut mettre deux heures pour faire quinze kilomètres sur la rocade. Vous comprendrez, madame la secrétaire d'État, qu'il y a véritablement urgence.

réponds au nom d'Élisabeth Borne, ministre chargé des transports, qui n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui. Le Gouvernement est sensible à la problématique de la congestion du trafic sur la rocade bordelaise, qui combine un trafic local, largement majoritaire, et un trafic de transit. Comme vous le soulignez, un grand contournement autoroutier avait été envisagé, voilà plus d'une dizaine d'années, afin d'écarter le trafic de transit de cet itinéraire. Il s'agissait d'une infrastructure autoroutière d'une centaine de kilomètres en tracé neuf, d'un coût estimé à plus de 1 milliard d'euros. Conformément aux orientations du Grenelle de l'environnement, ce projet a été abandonné en 2008. Il ne répondait pas à une nécessité de sécurité ou d'utilité collective et présentait un impact non négligeable sur l'environnement. De nouvelles propositions de contournement de Bordeaux ont été émises récemment par la métropole. Elles concernent la création d'un barreau autoroutier entre les autoroutes A62 et A89, à l'est du département de la Gironde. Elles sont actuellement étudiées par le Conseil d'orientation des infrastructures, qui est chargé, dans le cadre des assises de la mobilité, de proposer au Gouvernement une loi de programmation de nos infrastructures de transport, financièrement équilibrée, à un horizon de cinq ans. L'État est conscient des problèmes de congestion que rencontrent quotidiennement les usagers de la rocade bordelaise. C'est pourquoi, depuis 2009, il s'est fortement engagé aux côtés de la métropole pour son élargissement à deux fois trois voies, afin de la sécuriser et de diminuer les temps de parcours. Les résultats sont très positifs : les trafics sur la rocade ont été fluidifiés et les voiries urbaines délestées. Mais soyez assuré, monsieur le sénateur, que le Gouvernement restera vigilant s'agissant du traitement de ces noeuds de congestion routière

faille l'opposer à la nécessaire amélioration de l'existant, la réalisation du Grand Paris Express est très attendue par les Franciliens et les Franciliennes, d'où les inquiétudes légitimes qui émergent depuis quelques mois s'agissant des éventuels retards de calendrier ou d'une modification du tracé initial. Les derniers chiffrages de la Société du Grand Paris font état d'un surcoût d'environ 10 milliards d'euros, tandis qu'un rapport du préfet de région évoque des optimisations de dépenses : autant d'éléments faisant craindre aux élus locaux et aux habitants de certains tronçons puisse être abandonnée ou retardée, peut-être au profit d'autres, plus en lien avec les jeux Olympiques, par exemple. Certes, le Président de la République a coupé court à certains doutes, en annonçant récemment le maintien de la ligne 16 et sa réalisation pour 2024. C'est une bonne nouvelle pour les territoires concernés, qui en ont tant besoin, et j'espère qu'il ne les décevra pas. Mais qu'en est-il des autres lignes ?

telle ligne plutôt que telle autre : le Grand Paris Express est un schéma d'ensemble, conçu pour bien fonctionner une fois toutes les lignes réalisées. En ce sens, je rejoins la motion votée le 9 novembre dernier par le conseil d'administration Orbival, cette association qui rassemble des élus de toutes les sensibilités politiques, pour demander le maintien de tous les projets en cours, chacune et chacun ayant pour seul objectif le développement des transports publics. Le Gouvernement peut-il à présent préciser ses intentions sur le respect du calendrier et sur le maintien du tracé dans son intégralité, afin de lever toutes les incertitudes

la sénatrice, Mme Élisabeth Borne, ministre chargée des transports, n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui et m'a donc chargée de vous répondre.

pour maintenir l'Île-de-France dans les tout premiers rangs des métropoles mondiales et faciliter la mobilité quotidienne de l'ensemble des Franciliens. Le Président de la République l'a rappelé récemment : ni l'opportunité ni le schéma d'ensemble de ce projet ne sont remis en cause. D'importants travaux ont démarré depuis maintenant près de dix-huit mois. Le premier tunnelier entrera en action dès le début de l'année prochaine à Champigny-sur-Marne, dans votre département, madame la sénatrice.

D'autre part, des surcoûts très importants sont apparus, à cause notamment de la difficulté des travaux souterrains. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a chargé le préfet de région de faire un point précis sur le programme de réalisation du Grand Paris Express, en tenant compte de tous ces éléments. Le préfet a remis son rapport à la fin du mois de septembre et ses propositions sont en cours d'analyse. Le Gouvernement annoncera ses choix très prochainement, en vue de préserver au mieux les objectifs de ce projet essentiel pour l'Île-de-France, tout en retenant un calendrier techniquement réaliste et compatible avec la trajectoire de nos finances publiques.

Depuis le 1 juillet 2017 et l'inauguration en grande pompe de deux nouvelles lignes à grande vitesse, Rennes n'est plus qu'à 1 heure 25 de Paris et Bordeaux à 2 heures 04. Ces chiffres font rêver les Calvadosiens, qui, à l'inverse, ne peuvent que déplorer la vétusté des infrastructures et des matériels roulants de leur réseau ferré, ferré, obsolète et délabré. Il faut en effet toujours compter 1 heure 55, au mieux, pour effectuer le trajet entre Paris et Caen, alors que seulement 230 kilomètres séparent les deux villes. Si l'Atlantique se rapproche de la capitale, la Manche reste une zone non prioritaire, totalement transparente pour l'État et la SNCF. Au regard de ce triste constat, le souhait du Gouvernement de mettre en pause une vingtaine de projets d'infrastructures en cours, dont celui de la ligne nouvelle Paris-Normandie, la LNPN, ne peut que susciter l'inquiétude. Rapprochant la Normandie et l'Île-de-France, la LNPN se veut largement connectée au réseau ferroviaire existant. L'objectif n'est pas seulement de réduire les temps de parcours, mais aussi d'augmenter durablement la capacité des lignes, d'assurer une meilleure régularité et ponctualité des trains, que de renforcer la desserte des territoires, des villes et des ports. Au-delà du transport de passagers et de marchandises, c'est bien l'aménagement de la vallée de la Seine, de la baie de Seine et la politique maritime de la France qui se jouent ici. À cet égard, personne ne peut comprendre aujourd'hui, à l'heure où les grandes métropoles mondiales choisissent l'ouverture maritime, que la Normandie voie ses perspectives de développement freinées par un réseau ferré inadapté et vieillissant.

Autant dire que le projet est renvoyé aux calendes grecques ! C'est vraiment faire peu de cas des difficultés récurrentes rencontrées par les usagers des lignes ferroviaires normandes, comme ceux de la ligne Paris-Caen-Cherbourg, que je connais bien. Comme l'a admis en 2010 le président-directeur général de la SNCF, cet établissement public, et donc l'État, ont « une dette envers la Normandie ». Il est grand temps que cette région prenne toute sa place dans le réseau ferroviaire français. Madame la secrétaire d'État, à l'heure où se tiennent les assises nationales de la mobilité, censées déboucher sur une loi de programmation, pouvez-vous nous confirmer que la LNPN est toujours une priorité pour l'État ? La

Elle n'offre clairement pas aujourd'hui un niveau satisfaisant de qualité, en raison du trafic important qui perturbe souvent la partie de la ligne actuelle la plus proche de Paris. Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie vise à y remédier. Il en est actuellement au stade des études de définition. Des zones de passage préférentielles ont été proposées lors du comité de pilotage, réuni le 26 octobre dernier, pour les sections considérées comme prioritaires. Le Gouvernement se félicite du très large consensus qui ressort des travaux de cette instance. Toutefois, comme vous le rappelez, le Gouvernement a souhaité engager une démarche inédite pour le financement de nos infrastructures. La définition d'une loi de programmation, financièrement équilibrée à un horizon de cinq ans, permettra de donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs. Elle permettra aussi de faire face à l'impasse budgétaire actuelle de 10 milliards d'euros résultant d'engagements disproportionnés pris par le passé. Cette loi sera présentée au Parlement au premier semestre de 2018. Il s'agit d'une pause, et non d'une remise en cause du projet. Des propositions seront formulées par le Conseil d'orientation des infrastructures sur les grands projets ferroviaires. Nous recherchons déjà les solutions d'optimisation des réseaux afin de renforcer rapidement l'offre de service. C'est le sens des travaux engagés autour du complexe ferroviaire de Saint-Lazare, qui est déterminant pour la Normandie. Soyez donc assurée, madame la sénatrice, que le Gouvernement restera mobilisé pour apporter des réponses efficaces à une situation effectivement pénalisante pour des milliers d'usagers.

Forte de sa tradition maritime et de ses atouts en la matière, la Bretagne concourt à la formation de celles et ceux qui embrassent une carrière maritime. À cet égard, l'ENSM de Saint-Malo joue bien évidemment un rôle essentiel, au côté d'autres organismes. En décembre 2016, en partenariat avec l'ENSM, la région Bretagne, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo et la ville ont souhaité insuffler une nouvelle dynamique à l'école, en l'intégrant à un projet territorial moderne et réfléchi. Il s'agissait de délocaliser l'ENSM, présentement située au sein de la ville close, pour la rapprocher du lycée public maritime Florence-Arthaud. L'intérêt d'une telle opération réside notamment dans les mutualisations attendues entre l'ENSM et l'établissement du secondaire.

À terme, et d'un point de vue plus prospectif, un tel rapprochement peut enclencher un mouvement très favorable, à travers l'ouverture de nouveaux sites, dans le secteur de l'aéronautique en particulier, et être ainsi un premier pas vers la constitution d'un pôle maritime d'excellence. Puisqu'aujourd'hui, notamment depuis ce matin, nous savons la volonté du Gouvernement de permettre des rapprochements intelligents, j'aimerais cependant, madame la secrétaire d'État, que vous précisiez certains points quant à la concrétisation de ce projet territorial structurant sur le maritime mutualiser les fonctions supports entre l'école et le lycée public serait une bonne chose, mais pouvez-vous nous garantir que ce rapprochement maintiendra le haut niveau de qualification prodigué par l'ENSM et n'affectera pas

je vous réponds à la place de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui n'a pu être présente aujourd'hui. Je ne vais pas

quatre écoles historiques de la marine marchande, a prouvé, en sept ans d'existence, qu'elle pouvait moderniser ses enseignements et diversifier son offre de formation. Le résultat de ces efforts est tangible, puisque l'attractivité de l'école auprès des lycéens s'améliore et que le taux d'emploi des ingénieurs-navigants à la sortie de l'école est supérieur à la moyenne des grandes écoles. Le Gouvernement entend saisir l'occasion du nouveau contrat d'objectifs et de performance 2018-2020 pour franchir une nouvelle étape et affirmer l'ENSM comme une école maritime de référence à l'échelle tant nationale qu'internationale, en développant ses capacités pédagogiques, ses partenariats académiques et la recherche. Cette ambition passe par la poursuite du processus de rationalisation de l'établissement, aujourd'hui en surcapacité. L'éclatement de l'équipe de direction entre quatre sites nuit également au portage du projet de développement. Rechercher des économies sur les charges de structure ne signifie pas supprimer toute présence de l'ENSM à Saint-Malo ou à Nantes. Un travail est dans ce contexte engagé avec les acteurs des régions Bretagne et Pays de la Loire pour définir des projets qui permettront l'accueil de formations

terminé avec les réponses à des questions orales. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures

La séance est suspendue.